alors qu’il me revient de vous présenter les crédits du programme 161 « Sécurité civile », je ne peux commencer sans rendre hommage aux sapeurs pompiers, personnels navigants, formations militaires et associations agréées de sécurité civile, qui s’investissent sans compter dans la lutte contre les crises touchant notre pays chaque année. Grâce à leur engagement sans faille, la campagne de lutte contre les feux de forêt de l’été 2023 a pu être maîtrisée, après une année 2022 marquée par des incendies d’une ampleur exceptionnelle. Ces événements ont démontré la nécessité pour la sécurité civile de disposer de moyens à la hauteur de l’intensification et de l’extension géographique des différents risques induits par le changement climatique. À cet égard, l’on ne peut que se féliciter de l’augmentation des crédits du budget du programme 161, qui s’élèvent à 880,5 millions d’euros pour l’année 2024, soit une hausse d’un peu plus de 23 % par rapport à 2023.

afin de financer notamment la création d’une nouvelle unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, le renforcement des colonnes de renfort et le financement de nouveaux hélicoptères. Si je me félicite de l’augmentation des moyens consacrés à la sécurité civile, je regrette en revanche la méthode employée par le Gouvernement, qui, pour la deuxième année consécutive, a modifié substantiellement les crédits du programme 161 en cours de navette. Ce procédé n’est pas satisfaisant, car il nuit à la clarté des débats au Parlement. La méthode est d’autant plus contestable que l’amendement visait à financer des mesures annoncées par le Président de la République voilà un an. J’en viens maintenant aux nécessaires investissements dans les moyens aériens de la sécurité civile. Je me félicite de la concrétisation en 2024 du renouvellement de notre flotte d’hélicoptères Dragon. Près de 65,3 millions d’euros en crédits de paiement sont prévus pour l’année 2024, qui sera marquée par la livraison des trois premiers hélicoptères H145. Au total, trente six hélicoptères seront livrés d’ici à 2029, ce qui portera la flotte à quarante appareils. Je souhaiterais toutefois faire part à la Haute Assemblée de mon inquiétude concernant le renouvellement de notre flotte vieillissante de canadairs, qui tarde à se matérialiser. Une commande financée par l’Union européenne a, certes, été actée, et la France devrait bénéficier dans ce cadre de la livraison de deux canadairs, auxquels s’ajouteront probablement deux autres appareils financés sur fonds propres. Cependant, nous ne pouvons pas espérer acquérir le premier avion avant 2027, compte tenu des délais de production de ces appareils. Le Président de la République avait pourtant promis dans son discours du 28 octobre 2022 que la flotte de douze canadairs existants serait totalement renouvelée et portée à seize appareils d’ici à la fin de son quinquennat. Le Président de la République a également annoncé une commande de deux hélicoptères lourds bombardiers d’eau, dont la concrétisation se fait également attendre. L’intérêt opérationnel de ces appareils a largement été démontré, notamment lors de la saison des feux de forêt de Le ministère de l’intérieur a en effet eu recours à la location de dix hélicoptères de ce type, dans le cadre d’un marché de quatre ans, dont le coût annuel est estimé entre 16 millions d’euros je note que le PLF pour 2024 ne prévoit qu’une enveloppe de 7 millions d’euros consacrés à ces locations d’aéronefs. Je souhaiterais donc que Mme la ministre nous confirme que l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale permettra bien de couvrir l’ensemble des dépenses destinées à ces contrats de location. En tout état de cause, il me semble important que l’État puisse acquérir au plus vite ces appareils, qui – je le précise – ont vocation non pas à se substituer aux canadairs, mais plutôt à diversifier nos moyens de lutte contre les incendies. Le budget 2024 marquera également la poursuite de la mise en œuvre des pactes capacitaires, destinés à renforcer les moyens opérationnels des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) par l’acquisition de matériels cofinancés par l’État.

Si la première année de mise en œuvre de ces pactes capacitaires semble satisfaisante du point de vue de la plupart des Sdis, certains doutes subsistent quant aux délais de livraison des véhicules, compte tenu des difficultés rencontrées par les industriels sur les chaînes internationales d’approvisionnement. Le texte initial prévoyait une enveloppe de 7,4 millions d’euros en CP pour la poursuite de ces pactes capacitaires, renforcée à hauteur de 39 millions par l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale. Je m’en félicite, mais je regrette que nous ne disposions d’aucune visibilité sur l’échéancier d’exécution du reste des crédits destinés aux pactes capacitaires dans les prochaines années. Je conclurai mon propos en évoquant un projet qui me tient à cœur : le programme de mutualisation des systèmes d’information des Sdis, NexSIS 18 112. La fin de l’année 2023 est marquée par le déploiement effectif de NexSIS au sein des deux premiers Sdis. Une deuxième vague de déploiement devrait intervenir en 2024. Pour permettre la montée en puissance du projet, la subvention de l’État à l’Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) est portée cette année à 16,6 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 67,5 % par rapport à 2023.

Mes chers collègues, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose d’adopter les crédits de la mission « Sécurités ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec un budget de la gendarmerie en forte hausse, passant de 9,9 milliards d’euros à 10,4 milliards d’euros, la trajectoire de progression régulière fixée par la Lopmi est respectée. Il faut évidemment s’en féliciter. Ce budget finance notamment la création nette de 848 ETP, le déploiement des 239 nouvelles brigades, et la montée en puissance de la réserve opérationnelle,

En y ajoutant les effets de l’inflation, nous arrivons à un coût de près de 400 millions d’euros ! D’où un effet d’éviction massif pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement, à commencer par l’investissement immobilier, vrai sacrifié de ce budget, qui ne respecte la trajectoire de la Lopmi qu’en apparence.

il est indispensable de donner des instruments financiers pour faciliter le montage des projets. Sur ce point, les retours du terrain ne sont pas nécessairement positifs. Par exemple, les collectivités n’ont pas toujours la possibilité d’accorder des garanties d’emprunt aux opérateurs chargés de la construction.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l’a souligné mon corapporteur, ce budget de la gendarmerie, qui est en augmentation notable, respecte l’engagement pris dans le cadre de la loi de programmation.

que l’investissement immobilier, le renouvellement de la flotte de véhicules légers est en panne, avec seulement 500 véhicules acquis, alors que 3 700 seraient nécessaires pour rajeunir le parc. Après les années favorables de 2020 à 2022, nous sommes clairement revenus à une tendance baissière qui ne pourra pas perdurer. une bonne nouvelle : l’arrivée des cinquante huit derniers blindés Centaure, qui remplacent progressivement les vieux véhicules à roues de la gendarmerie, mis en service en 1974. Les dépenses de fonctionnement demeurent stables, ce qui, compte tenu de l’inflation, constitue une baisse en valeur. Le fonctionnement courant lié à l’agent est ainsi en diminution de 19,4 %. Presque tous les postes sont affectés : la baisse des dépenses de formation, à –35 %, n’envoie pas un bon signal alors que la gendarmerie a l’ambition de recruter massivement et que ses missions évoluent. De même, les dépenses de fonctionnement liées aux moyens mobiles sont particulièrement touchées, alors que les effectifs s’accroissent, en contradiction avec la doctrine de « l’aller vers ». Avec ces coups de rabot, nous sommes loin de la logique vertueuse de programmation pluriannuelle, comme l’a souligné la Cour des comptes. Je terminerai mon propos en évoquant l’emploi de la réserve opérationnelle. L’appui de la réserve sera indispensable au cours de l’année 2024, lors de laquelle 12 000 à 14 000 gendarmes devraient être mobilisés sur une courte période à l’occasion des jeux Olympiques. Mais dans quelles conditions les renforts seront ils mobilisés et les réserves employées ? La perspective risque d’être peu motivante, au vu des difficultés de logement caractéristiques de la région parisienne, qui seront amplifiées par l’événement. L’audition du directeur général de la gendarmerie nationale par notre commission n’a pas permis de lever toutes les incertitudes. Cette question dépasse les échéances de court terme. Entre les événements exceptionnels, les catastrophes naturelles qui se multiplient et des formes de contestation de plus en plus difficiles à maîtriser, les gendarmes ont parfois le sentiment de ne plus pouvoir assumer leurs missions du quotidien. À l’heure où tous les corps militaires sont confrontés à des difficultés de recrutement et de fidélisation, il est indispensable de s’assurer que les jeunes gendarmes comprennent le sens de leur mission et ne doutent pas de disposer des moyens de la remplir pleinement. Je formulerai, à l’instar de mon corapporteur et de notre commission, un avis favorable sur l’adoption des crédits de ce programme : ne pas voter des crédits en augmentation marquerait un manque de soutien à notre gendarmerie. Mais la soutenir, c’est aussi lui donner à l’avenir tous les moyens d’exercer pleinement l’ensemble de ses missions. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des lois a émis un avis favorable sur l’adoption des crédits de la mission « Sécurités ». Il me revient de vous les présenter au nom de notre collègue Henri Leroy. Ce projet de loi de finances est en effet globalement conforme à la programmation adoptée par le Parlement dans le cadre de la Lopmi. IL va donc dans le bon sens, car il permet de mettre en œuvre pour la deuxième année une programmation conforme aux besoins et aux attentes tant des forces de l’ordre de nos concitoyens en matière de sécurité. La commission a toutefois assorti de quatre principales réserves son avis favorable sur l’adoption des crédits. La première est due, dans l’exécution des budgets 2023 et 2024, aux effets de l’inflation. La Lopmi a été élaborée avant la survenue de ce phénomène, qui n’a pas conduit à revaloriser les budgets décidés. La police et la gendarmerie nationales vont donc devoir participer à l’effort national de rationalisation des dépenses, mais cela ne devra pas porter préjudice à la capacité des forces à faire face aux échéances de 2023 et 2024. La deuxième tient au fait que l’exercice 2024 sera particulier pour les forces de sécurité intérieure, compte tenu des importants défis organisationnels et sécuritaires qui devront être relevés, s’agissant en particulier de l’organisation et de la sécurisation des jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et sur trente Toutefois, nous ne sommes pas aujourd’hui en mesure d’estimer le coût de sécurisation de ces jeux, ce qui, compte tenu des difficultés de pilotage des dépenses, constitue inéluctablement un facteur de tension sur les crédits alloués aux deux forces, particulièrement en fin de gestion. La troisième réserve porte sur la nécessaire diminution de la part des dépenses de personnel dans les dépenses totales de ces deux programmes. Une telle dépendance à la sous consommation des crédits de personnels n’est pas souhaitable. Une évolution structurelle est nécessaire, et la commission des lois s’y montrera attentive. Enfin, notre dernière réserve porte sur l’évolution divergente des crédits titre 2 entre les deux forces, qui sont pourtant confrontées à des difficultés similaires et à une surcharge d’activité du même ordre. Un tel décrochage ne peut être que temporaire et doit faire l’objet de mesures de rééquilibrage dès l’année prochaine au profit de la gendarmerie nationale ; nous y serons vigilants.

de la sécurité civile. Nous saluons la continuation des efforts engagés depuis l’année dernière, afin de soutenir les services d’incendie et de secours et de procéder au renforcement de la flotte aérienne de la sécurité civile. Les terribles incendies de l’année 2022 auront au moins permis une salutaire prise de conscience quant à la nécessité d’adapter nos moyens de lutte contre les incendies de forêt aux défis qu’engendre le changement climatique. Cette année encore, malgré un été pluvieux sur une large partie du territoire – cela a permis de contenir le nombre d’hectares brûlés dans la moyenne des vingt dernières années –, nous avons observé une extension de la période des feux, qui apparaît moins cantonnée aux seuls mois de juillet et d’août. Nous assistons donc depuis plusieurs années à une transformation des risques, qui exige des réponses. Je souhaite rappeler à ce titre que le Sénat est particulièrement mobilisé pour accompagner tous les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’incendie, comme l’illustre notamment la promulgation récente de la loi, d’initiative sénatoriale, du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. C’est avec le même esprit de vigilance constructive que la commission des lois a abordé les crédits du programme 161 pour l’année 2024, qui affichent un maintien des autorisations d’engagement à un niveau élevé et une hausse significative des crédits de paiement. Nous nous réjouissons de la bonne avancée du renouvellement et de l’extension de la flotte d’hélicoptères H145, de l’accélération du programme NexSIS 18 112, qui va être déployé dans vingt départements l’année prochaine, ou encore de l’engagement de nouveaux crédits de paiement consacrés aux pactes capacitaires, qui permettront de soutenir les services d’incendie et de secours, afin de renforcer leur flotte de camions citernes. Cette satisfaction est néanmoins obérée par plusieurs vives préoccupations. En témoignent les deux amendements que nous avons déposés, concernant, l’un, l’engagement présidentiel de doter la France de deux hélicoptères lourds, l’autre, le calendrier de consommation des crédits dédiés aux pactes capacitaires. J’y reviendrai lors de la discussion des amendements. Outre ces deux points, nous regrettons en particulier l’opacité qui caractérise la commande des seize nouveaux canadairs. Nous comprenons qu’il existe des difficultés de production liées à la situation monopolistique du constructeur. convient cependant que la parole publique, en particulier celle du Président de la République, soit suivie d’effets et que les éventuelles difficultés soient recensées avec transparence. À ce titre, nous appelons à la mise en œuvre intégrale des annonces du Président de la République du 28 octobre 2022, incluant aussi bien le plan d’extension de la flotte que le plan de renouvellement des douze appareils actuels. Mes chers Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de quinze minutes pour intervenir. Dans la suite

Tant de violences ont émaillé l’année qui s’achève, pendant laquelle nos forces de sécurité ont été mises à rude épreuve. En plus d’assurer la sécurité au quotidien, les forces de l’ordre doivent protéger nos concitoyens contre la menace djihadiste

notamment irréguliers. Surveiller les frontières et éloigner les étrangers qui doivent quitter notre territoire sont deux missions qui requièrent de plus en plus de personnel.

Ensuite, il renforce la présence policière sur le terrain, ce qui est fondamental pour nos concitoyens. La Lopmi prévoit ainsi la création de 200 brigades de gendarmerie et de onze unités de force mobile, et nous visons toujours l’objectif de création de 8 500 postes de policiers et gendarmes d’ici à 2027. L’emploi de la réserve opérationnelle implique aussi que celle ci dispose de locaux et de matériels. Il faut que l’intendance suive. Ce budget le prévoit. Enfin, le développement technologique rend essentiel l’achèvement du déploiement du numérique au sein de nos forces. Ce budget l’acte. À ces questions

à la sécurité routière. Ensuite, les crédits que nous examinons doivent nous permettre de lutter contre les conséquences les plus immédiates du dérèglement climatique. Les départements du nord de la France sont confrontés à des inondations d’ampleur depuis de longues semaines. Chaque année, les feux de forêt font partir des centaines d’hectares en fumée. La réduction des surfaces brûlées, qu’il faut souligner, montre l’efficacité de nos services, mais l’accroissement du nombre de départs de feux rend leur mission de plus en plus difficile ; il faut en tenir compte.

Ce budget prévoit le renforcement des effectifs des réserves opérationnelles des deux forces, la création de 8 500 postes et, enfin, l’instauration de 200 nouvelles brigades de gendarmerie et de 11 nouvelles unités de force mobile.

Ensuite – vous connaissez mon penchant pour le sujet –, j’espère que ce budget sera également l’occasion d’une poursuite des efforts dans le traitement des violences intrafamiliales l’occurrence, nos policiers et nos gendarmes sont en première ligne. Un dépôt de plainte n’est jamais un moment agréable, quel qu’en soit le motif, mais pour une victime de violences conjugales, c’est un moment particulier, un instant de bascule,

Certes, madame la ministre, je reconnais bien volontiers les efforts de ces dernières années. Mais ils sont inégalement répartis sur le territoire et une victime joue à la roulette russe : tout peut très bien se passer si elle tombe sur un policier formé, elle peut être renvoyée à sa triste condition avec un policier qui ne l’est pas. Les formations doivent donc se poursuivre. Je souhaite également insister sur le besoin de généraliser le recours aux intervenants sociaux en gendarmerie et en commissariat.

Si l’on tient compte de l’inflation et d’une modification du périmètre de la mission, les moyens pour la sécurité civile diminuent. L’adoption d’un amendement du Gouvernement, déposé à l’Assemblée nationale, permet tout juste de financer l’achat de nouveaux camions citernes, de renouveler la flotte des hélicoptères et de créer une nouvelle unité d’intervention et d’instruction.

infrastructures en élargissant les digues ou en renouvelant les wateringues, qui servent à évacuer l’eau plus rapidement vers la mer. D’autre part, il faudrait aussi recruter et investir dans les moyens techniques de la protection civile, par exemple pour acheter des engins de pompage.

plus de formation. Cet été, la Cour des comptes a rappelé les capacités limitées des écoles de police et a alerté précisément sur le fait que même des recrutements massifs ne permettent pas de résoudre des « difficultés structurelles

peuvent être très positives – et les dispositifs spécifiques qui existent déjà, ici ou là, ne pourront guère porter leurs fruits. Je salue les 260 intervenantes et intervenants sociaux dans les commissariats ou les 99 nouvelles maisons de protection des familles pour aider les victimes de violences intrafamiliales. Mais aussi longtemps que

par l’existence d’une force publique « instituée pour l’avantage de tous » ; celle ci doit être correctement financée. Ainsi, et notre groupe en est convaincu, l’aspiration à la sécurité doit être une priorité, au même titre que le combat pour la santé, pour le logement ou pour les transports. Et l’action des fonctionnaires les font vivre au quotidien doit être saluée. C’est pourquoi nous pensons que les moyens alloués à la police et à la gendarmerie nationales dans ce projet de loi de finances ne sont malheureusement pas à la hauteur des attentes des citoyens en matière de liberté et de tranquillité.

Nous avons tous en tête la note publiée au mois de juillet dernier par la Cour des comptes, selon laquelle la progression des crédits prévue dans la Lopmi « ne règle pas les difficultés structurelles des forces de sécurité intérieure ». ». Ces dernières rencontrent des difficultés croissantes de recrutement et une nette augmentation des départs et des démissions. En 2022, on a déploré 10 000 départs de policiers et 15 000 départs de gendarmes. outre, la Cour des comptes met en évidence que les fortes ambitions affichées sur l’équipement et l’investissement ne trouvent pas de traduction suffisante dans la programmation. J’ajoute, à l’instar de ma collègue Mélanie Vogel, que les lacunes en matière de formation Le nombre d’heures de formation est annoncé comme étant « en hausse », mais le tableau présentant les éléments de synthèse du programme affiche des zéros dans la colonne des dépenses de personnel. Autrement dit, les promesses d’une meilleure formation pour nos policiers, dont le nombre augmente, ne se traduisent par aucun investissement concret. Pourtant, les agents sont unanimes à demander des formations, notamment en matière de tir,

Nous déplorons par ailleurs que l’essentiel de ces crédits soit consacré à la vidéosurveillance. Nous croyons qu’il est primordial de s’attaquer aux causes et non aux seules conséquences, en privilégiant la prévention et la dissuasion. Ce qui nous préoccupe le plus, c’est la persistance d’une grande souffrance au travail, qui nous presse d’améliorer significativement les conditions de travail des policiers et des gendarmes. Depuis vingt ans, nous comptons plus de mille suicides parmi nos policiers. Chaque fois que l’on renonce à lutter contre ces suicides, chaque fois que l’on ne consacre pas de moyens à l’aide psychologique des agents qui en font la demande, c’est la démocratie qu’on abîme, c’est tout notre système qu’on empêche de fonctionner correctement. Les crédits du programme 161 « Sécurité civile » n’augmentent que de 2,87 %, alors que le dérèglement climatique est à l’origine de catastrophes majeures. Cette augmentation nous paraît insuffisante. Il y a quelques jours, notre pays a connu des tempêtes équivalentes à celles de 1999.

ont mis en évidence le manque structurel d’effectifs de sapeurs pompiers. Les sapeurs pompiers et les présidents de département n’ont plus les moyens de faire face à la progression du nombre d’interventions.

lutte contre le terrorisme, contre la délinquance quotidienne, contre la cybercriminalité ou encore contre les feux de forêt… voilà donc une mission aux enjeux hétérogènes, mais sûrement pas hétéroclites Ces différentes actions n’ont finalement qu’un seul objet : garantir la sûreté dans notre Nation, ce qui constitue le préalable pour une société qui aspire à une vie paisible. Le discours sur la sécurité est trop souvent l’objet de préjugés ou de confiscations par une partie de la classe politique. C’est un tort : l’État doit être le gardien de la liberté individuelle de chacun. Et pour y parvenir, il est nécessaire qu’un nombre suffisant de femmes et d’hommes se mobilisent et se dévouent pour garantir la sécurité quotidienne de nos concitoyens. Aussi, je vais partir d’une observation simple sur ce PLF pour 2024 : le budget alloué à la police nationale est en hausse, tout comme celui de la gendarmerie nationale ; cela nous convient. Bien entendu, une telle augmentation était attendue après l’adoption de la Lopmi, qui intervient dans un contexte d’extrême sollicitation des forces de l’ordre, notamment dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques de 2024. Nous la saluons, d’autant plus que nous sortons de l’organisation de la Coupe du monde de rugby, qui, si elle ne s’est pas traduite par une victoire de nos Bleus sur le terrain,… À notre grand regret ! … aura été un succès certain en matière de sécurité publique.

Réjouissons nous que notre pays demeure capable d’accueillir de tels événements mondiaux ! Il ne reste plus qu’à espérer que cela se poursuive ainsi lors des jeux Olympiques et Paralympiques l’été prochain. Il est donc prévu de renforcer les effectifs, notamment le recrutement de nouvelles unités de force mobile, spécialisées dans la sécurisation des grands événements, ou encore d’augmenter ceux des réserves opérationnelles.

les réseaux de formation sont sous pression constante depuis dix ans, notamment du fait de la réduction des infrastructures et de l’augmentation des recrutements et des besoins de formation. moyens s’ajoutent d’autres carences. D’un côté, la formation initiale est confrontée à une baisse du niveau des élèves. De l’autre, la formation continue n’est pas suffisamment rapprochée des besoins des équipes de terrain.

–, s’il est nécessaire d’augmenter le nombre d’agents pour répondre au surmenage des services, cette augmentation doit être accompagnée d’un gage de qualité

permettant à l’État d’assurer ses fonctions ont été fortement négligées par les majorités qui se sont succédé depuis une trentaine d’années. Nos armées ont été budgétairement asphyxiées, et leurs capacités opérationnelles considérablement réduites. Les conditions d’exercice de la justice n’étaient pas dignes d’un grand pays comme le nôtre. Nos forces de sécurités intérieures, quant à elles, ont été confrontées à une carence en moyens humains et matériels, que seul un engagement exceptionnel des policiers et des militaires de la gendarmerie est venu en partie compenser, alors même que les tensions au sein de la société étaient déjà grandissantes. Enfin, les défis représentés par l’évolution des risques liés à sécurité civile liés au changement climatique n’étaient tout simplement pas pris en compte. Ce quinquennat sera celui de la reprise en main par l’État

Au total, ce quinquennat sera celui de la restauration de la capacité de l’État à asseoir son autorité, dans un contexte que nous savons de plus en plus complexe. En ce qui concerne plus particulièrement les crédits de la mission « Sécurités nous constatons avec satisfaction que, pour la deuxième année consécutive, les engagements pris par la Gouvernement dans le cadre de la Lopmi trouvent leur traduction budgétaire, en espèces sonnantes et trébuchantes, dans le PLF.

création de 1 139 emplois dans la police nationale et de 1 045 emplois dans la gendarmerie. Ces moyens supplémentaires permettront de mieux assurer la sécurité de nos concitoyens. Permettez moi de me réjouir tout spécialement de la création de 239 brigades de gendarmerie, qui viennent conforter le maillage territorial, essentiellement ces nouvelles brigades va toutefois remettre en perspective la politique immobilière de la gendarmerie. À cet égard, le système en vigueur actuellement n’est pas satisfaisant. Les collectivités locales sont en effet beaucoup trop sollicitées pour ce qui relève d’une compétence régalienne. Sans même évoquer le contexte inflationniste, les évolutions décidées par l’État des normes sécuritaires et environnementales ont considérablement renchéri les coûts des projets de caserne. Aussi, les collectivités doivent de plus en plus mettre la main à la poche. Pour faire passer la pilule, et parce que les loyers versés par l’État central sont bien souvent insuffisants pour couvrir les annuités des emprunts contractés, l’État local se voit de plus en plus fréquemment contraint de soutenir également les collectivités dans ces projets immobiliers

Mme la rapporteure pour avis Françoise Dumont, dont je tiens à saluer la qualité du travail, a d’ailleurs souligné que les crédits de paiement avaient augmenté de 76 % par rapport à la moyenne de la précédente décennie.

Nous savons cependant que 80 % des sommes dédiées à la sécurité civile le sont par les services départementaux d’incendie et de secours, qui sont essentiellement financés par les collectivités. Certes, l’État est venu concrètement à leur soutien, au moyen du pacte capacitaire. Mais il faudra nécessairement revoir les modalités de leur engagement dans les années à venir. Osons le dire : certains Sdis sont aujourd’hui sous financés ; d’autres doivent encore prendre toute la mesure des évolutions à conforter ! Ainsi, l’évolution des risques doit également conduire, outre les seules questions opérationnelles, à une réforme du financement des Sdis, dont les enjeux financiers seront d’une tout autre ampleur. La mission « Sécurités » du PLF 2024 apporte donc de très nombreuses satisfactions. Nous sommes convaincus que les budgets alloués permettront de faire face aux besoins. Cependant,

Quelle que soit la qualité du travail de prévision budgétaire, celui ci ne peut évidemment pas anticiper tous les besoins qui se font jour au fur et à mesure de l’avancement de l’organisation de l’événement.

La capacité de l’outil industriel à répondre aux commandes est au cœur des préoccupations de la sécurité civile. Nous pouvons le constater aujourd’hui dans la mise en œuvre du pacte capacitaire avec des délais de livraison des matériels, pourtant financés et commandés, qui s’allongent terriblement. Nous l’observons également à propos des moyens aériens. Je pense en particulier aux canadairs, dont la chaîne de production est à l’arrêt depuis maintenant de nombreuses années. Dans un contexte mondial de reprise extrêmement forte des commandes d’aéronefs civils,

Si tout ne nous allait pas dans ce texte, il nous semblait juste et utile de soutenir une politique budgétaire assumant une hausse des moyens consacrés à la sécurité. Ce vote ne valait pas pour nous quitus sur l’ensemble de nos différends avec le Gouvernement qui, s’il était besoin de le préciser, Cette Lopmi sous tendait des hausses d’effectifs. Les créations de postes se poursuivront en 2024 avec l’annonce de 2 184 policiers et gendarmes supplémentaires. Pourtant, le diable se cache dans les détails.

d’un “recrutement massif de policiers et de gendarmes”, les responsables de programme sont contraints de dégrader la qualité des recrutements et des formations, d’autant que les viviers de recrutement s’assèchent peu à peu. » les forces de l’ordre entrent en concurrence avec d’autres recruteurs, comme les polices municipales, les sapeurs pompiers, la sécurité privée et les forces armées, dont les effectifs et agents sont également amenés à croître dans les prochaines années. À titre d’exemple, la même Cour des comptes, dans une note du mois de novembre 2021, de 2014 à 2020, le taux d’admission au concours de gardien de la paix était passé de 2 % à 18 % des candidats, tandis que les formations de gardien de la paix et d’officier avaient été raccourcies. S’agissant de la formation, justement, le projet de loi de finances soulève des interrogations sur la réalité des moyens alloués, comme d’autres orateurs l’ont souligné. Un des objectifs de la Lopmi est d’augmenter de 50 % le temps de formation continue des policiers. Les indicateurs présentés dans les documents budgétaires font plutôt état d’une légère dégradation de l’effort de formation, puisque, de 2021 à 2022, le nombre d’heures de formation continue individuelle ou collective par actif est en diminution : 31,20 heures en 2021, 30,90 heures sur l’année 2022. Pour inverser cette tendance et atteindre les objectifs fixés par la Lopmi, des moyens supplémentaires devront être mobilisés. Or les dépenses de formation du programme « Police nationale » connaissent une forte baisse

Interpellé à ce sujet lors de son audition par la commission des lois de l’Assemblée nationale, le ministre Darmanin a contesté ces chiffres, affirmant : « Les crédits de formation en personnel ne baissent pas – soit il y a des coquilles dans le document budgétaire, soit il faudra le relire ensemble : ils sont passés de 23 millions en 2022 à 29 millions en 2023 et seront de 30 millions l’année prochaine, avec 4 500 équivalents temps plein et 72 ETP recrutés et créés, en sus des policiers qui basculent dans la formation. » Si le chiffre pour 2024 est bien exact, soit 29,7 millions d’euros pour être précis,

les documents budgétaires pour 2024 n’évoquent pas ces soixante douze ETP. Sur ces deux points, des éclaircissements de Mme la ministre seraient bienvenus ! À propos de cette mission « Sécurités », il convient de rappeler l’implication de la commission des affaires étrangères dans l’examen des crédits de la gendarmerie nationale. Ce programme est suivi par deux corapporteurs, Philippe Paul et Jérôme Darras, que je salue. Sur cette question, les crédits de la mission semblent bien s’inscrire dans la trajectoire de la Lopmi, sous réserve d’évoquer plusieurs points de vigilance. En effet, l’accroissement des dépenses de personnel du titre 2, dont nous pouvons nous satisfaire, se fera au détriment des dépenses de fonctionnement et d’investissement. L’immobilier était déjà un enjeu crucial pour la gendarmerie. Or les problèmes seront accentués par les besoins de logement des nouvelles brigades, fixes et mobiles, par les collectivités d’accueil. Par exemple, dans mon département, les solutions reposent beaucoup sur la bonne volonté du conseil départemental, même si le sujet dépasse ses compétences.

orateurs l’ont signalé. Par conséquent, si l’immobilier se trouve de plus en plus maltraité et si les équipements, notamment les véhicules, ne suivent pas, nous en arriverons paradoxalement à annuler les effets attendus des revalorisations indemnitaires et des recrutements des gendarmes. Cette mission contient également le programme « Sécurité civile

au printemps 2024. Après quelque 70 millions d’euros en 2023, ce sont 66 millions d’euros qui sont inscrits au budget 2024 pour financer le renouvellement de la flotte. Le groupe socialiste appelle cependant de ses vœux à un effort budgétaire supplémentaire pour accroître le soutien aux Sdis,

Des syndicats de policiers se font très pressants envers le ministère, certains évoquant même un ultimatum. Au delà de ce climat social, qui fait couler beaucoup d’encre, cela soulève quelques questions s’agissant de la sincérité du budget proposé.

cela a déjà été dit, les crédits pour 2024 de la mission « Sécurités » connaîtront une croissance de 1,16 milliard d’euros en autorisations d’engagement et de 1,04 milliard en crédits de paiement, représentant une progression de l’ordre de 5 % de la dotation en crédits de paiement de chacune des forces. des forces. Pour la deuxième année de mise en œuvre de la Lopmi, nous saluons la conformité globale des crédits à la programmation adoptés par le Parlement le 24 janvier dernier. Les moyens alloués à ceux qui nous protègent doivent être à la hauteur de l’exigence et de la difficulté de leur mission au service de nos concitoyens. Toutefois, à la lumière de l’exécution du budget pour 2023, les pistes d’économies suggérées par la Cour des comptes nous semblent insuffisamment prises en compte. Ainsi en est il de la répartition des zones police et gendarmerie. À l’instar de la Cour, nous regrettons que la mutualisation des moyens entre police et gendarmerie ne soit pas assez aboutie, notamment en ce qui concerne les logiciels de rédaction des procédures, la police technique et scientifique ou encore la cybercriminalité, où l’on recense un certain nombre de doublons. De même, l’action des forces de police et de gendarmerie doit se concentrer sur les formes les plus graves de criminalité et d’atteinte à l’ordre public, sans préjudice d’une meilleure association des quelque 35 000 agents de police municipale, dont le rôle est, au fil du temps, devenu fondamental. Nous sommes également très favorables au fait de privilégier des leviers non salariaux

Il y aura un après jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en péril la sécurité des Français à leur issue ! Il nous semble donc indispensable de mettre l’accent sur des mesures d’économies, dans un contexte inflationniste aigu qui pèse sur les dépenses de fonctionnement du ministère de l’intérieur. Je pense notamment à l’important coût de l’essence et de l’énergie. Par ailleurs, des inquiétudes légitimes, nous semble t il, demeurent quant au contexte sécuritaire inédit de l’année qui s’annonce ; cela a été relevé. À cet égard, nous souhaiterions savoir, madame la ministre, à quel coût le Gouvernement estime la sécurisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans un autre registre, la recrudescence des incendies en période estivale nous inquiète également, puisque, comme le soulignait notre collègue rapporteure pour avis Françoise Dumont de lourdes interrogations demeurent quant au calendrier de livraison des futurs canadairs, au regard des capacités de la chaîne de production canadienne, qui est à l’arrêt. Si les moyens aériens légers ont été renforcés, il ne faut pas oublier que la France a été forcée ces dernières années de recourir à la location au travers des sociétés privées, et ce à des conditions tarifaires peu favorables. Mes chers collègues, les nombreux défis qui se profilent nous obligent à faire preuve de responsabilité. C’est pourquoi je ne doute pas que la grande majorité de notre groupe votera en faveur de l’adoption des crédits de la mission « Sécurités » pour 2024. Je terminerai en remerciant chaleureusement nos rapporteurs spéciaux, Bruno Belin et Jean Pierre Vogel, ainsi que nos rapporteurs pour avis, Françoise Dumont, Henri Leroy, malheureusement empêché ce soir pour des raisons de santé, Philippe Paul et Jérôme Darras, de la qualité de leur travail. Chacun a su

de chiffre d’affaires : trafic de migrants, travail forcé, trafic aux fins d’exploitation sexuelle et d’activités criminelles contraintes… Parmi les dix priorités annoncées le 26 mai 2021 par le Conseil européen,

Je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser le ministre de l’intérieur et des outre mer, qui ne peut malheureusement pas être présent aujourd’hui, étant à l’Assemblée nationale pour défendre le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, texte que vous avez adopté le 14 novembre dernier. Dans le contexte que nous connaissons, mon intervention revêt un caractère singulier : jamais les Français n’ont autant eu besoin de sécurité et jamais l’État n’a mis autant de moyens au service de leur sécurité. Aussi, derrière les données budgétaires, ce sont bien des femmes et des hommes qui concourent à maintenir, dans des conditions parfois difficiles, l’ordre et la sécurité publique. Je leur adresse toute ma reconnaissance. Grâce à vous, l’année 2023 a été marquée par l’adoption de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, qui consacre près de 15 milliards d’euros sur cinq ans à la sécurité des Français. Je le répète devant vous : ces crédits doivent être exécutés conformément à la trajectoire budgétaire que vous avez votée. Si l’inflation et la prise sous plafond de mesures de revalorisation du point d’indice conduisent à des arbitrages internes au ministère, nos priorités demeurent inchangées demeurent inchangées : renforcer la présence des forces de sécurité intérieure sur la voie publique, lutter contre le terrorisme, affermir l’administration territoriale et préparer les jeux Olympiques et Paralympiques. Face aux menaces diverses, mais multiples, nous menons un effort sans précédent pour renforcer la présence des forces de sécurité intérieure (FSI) sur la voie publique, partout sur le territoire. Nous avons doublé la présence d’agents sur la voie publique, notamment par la fin des gardes statiques et par la substitution du personnel actif par du personnel administratif : 2 850 FSI nouvelles ont été déployées en 2023,

de notre présence passe aussi par un affermissement de l’ancrage territorial, par la création des 239 brigades territoriales sur cinq ans, en concertation avec les élus. fixes, 145 mobiles, dont 80 créées sur les annuités 2023 et 2024 pour un total de 690 ETP. Permettez moi de souligner que les brigades mobiles ont pour objectif de rapprocher les services de la brigade de gendarmerie des populations et de parcourir le dernier kilomètre. Certaines seront d’ailleurs thématisées. Il s’agit d’une action totalement inédite depuis la création de la gendarmerie nationale un effort particulier est prévu pour les outre mer. Il est nécessaire pour répondre aux enjeux de sécurité dans ces territoires et renforcer les moyens de lutte contre la délinquance et contre les stupéfiants en Guyane, de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte et contre les trafics illicites à la Martinique. Entre 2017 et aujourd’hui, ce sont 1 400 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été affectés dans ces territoires,

à la Guadeloupe et dans les îles du Nord, une à la Martinique, une à La Réunion et une en Polynésie. Cette dynamique de renforcement se poursuivra avec la création prochaine de vingt deux nouvelles brigades de gendarmerie, dont huit entre 2023 et 2024. En plus de la présence sur le terrain, les FSI ont connu un renforcement en matière d’équipements – vous avez été nombreux à le souligner –, afin de les accompagner dans leurs missions. Quelque 4 800 véhicules légers pour la police nationale et la gendarmerie nationale ont été acquis en 2023, après l’achat de 13 310 autres sur les deux dernières années. Depuis l’entrée en fonction de Gérald Darmanin, plus de la moitié du parc automobile a été renouvelée et le ministère fera l’acquisition de 3 600 nouveaux véhicules en 2024 pour 130 millions d’euros.

monsieur le rapporteur spécial Vogel, dans la continuité des annonces du Président de la République, le Gouvernement a déposé un amendement important concernant le renforcement des moyens consacrés à la sécurité civile, notamment pour lutter contre les feux de forêt, à hauteur de 140 millions d’euros en

mais aussi 39 millions d’euros au titre des pactes capacitaires, 32 millions d’euros pour les canadairs et 23 millions d’euros pour la location de moyens aériens, avions et hélicoptères bombardiers d’eau. Parallèlement, la fin de l’année 2023 verra la notification du marché visant à acquérir près de quarante nouveaux hélicoptères pour la sécurité civile et pour la gendarmerie nationale, pour un engagement de plus de 500 millions d’euros. C’est un effort important face à la recrudescence des incendies, dans un contexte de changement climatique et d’aggravation de la menace. Enfin, des ressources supplémentaires sont requises pour mieux répondre à la cybercriminalité, nouvelle frontière de la délinquance 1 500 cyberpatrouilleurs ont été recrutés, soit une hausse de 50 % par rapport à l’existant, et un appel d’urgence numérique, le « 17 cyber », a été mis en place. En outre, dans le cadre du plan France Ruralités, nous prévoyons des actions de sensibilisation auprès des communes et des maires, parmi les premières victimes de ces nouvelles menaces.

nous mettrons en effet en place la visioplainte et le portail Ma sécurité, afin d’accompagner, là encore, le dernier kilomètre des politiques publiques en matière de sécurité.

La Coupe du monde de rugby n’a donné lieu à aucun incident de sécurité grâce à une présence policière et militaire sans précédent. Les préfets ont mené, à la demande de Gérald Darmanin, près 4 800 opérations zéro délinquance, conduisant à 781 interpellations et à 475 gardes à vue. Par ailleurs, six drones ont été interceptés. Ces jeux constituent un événement hors norme trente sites, 206 nations représentées, 10 500 athlètes, trente deux sports, 329 épreuves et environ 10 millions de spectateurs cumulés attendus en Île de France.

hors hébergement, les conventionnements étant en cours, et hors gratifications qui pourraient être mobilisées. Un dispositif ministériel d’envergure définira une manœuvre de sécurité conçue et conduite au niveau national en renforçant la coordination entre les FSI,

: augmentation des crédits des plans départementaux d’action de sécurité routière, renforcement des partenariats associatifs et prévention outre mer.

du régime de la concession de logement par nécessité absolue de service inhérent au statut des officiers et des sous officiers de gendarmerie. Vous avez été nombreux à appeler une telle

: La parole est à Mme Marianne Margaté. lisant les différents documents budgétaires, il est frappant de constater que la taille de notre flotte aérienne de sécurité civile est semblable à ce qu’elle était voilà une trentaine d’années, alors que le contexte a considérablement évolué depuis lors ; nous le savons tous. Avec le changement climatique, les risques d’incendie se multiplient aussi bien dans l’espace que dans le temps. De plus, comme le souligne le rapport d’information sénatorial du mois de juillet dernier sur le sujet, le renouvellement de la flotte de bombardiers d’eau souffre d’un défaut d’anticipation.

Leur acquisition à l’unité est estimée par le rapport précité à 25 millions d’euros l’unité. Nous proposons donc des crédits supplémentaires à hauteur de 250 millions d’euros et nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

rapporteure pour avis. Cet amendement, que je présente au nom de la commission des lois, a pour objet de donner suite aux engagements formulés par le Président de la République lors de son discours aux acteurs de la lutte contre les feux de forêt,

la gestion des crises (DGSCGC) s’est montrée très évasive à chaque fois que je l’ai interrogée sur le sujet. Tout au plus m’a t on parlé d’un appel à projets européen ne portant que sur un seul hélicoptère lourd. En revanche, le recours à la location d’hélicoptères lourds, fort coûteux, s’est systématisé, puisqu’un marché pluriannuel pouvant atteindre jusqu’à 120 millions d’euros sur quatre ans a été signé récemment. Le coût unitaire d’un hélicoptère lourd H 225 est estimé à 46 millions d’euros,

d’envisager la concrétisation d’une commande de dix hélicoptères lourds, d’autant que les délais de fabrication de ces appareils et de construction des infrastructures susceptibles de les accueillir peuvent atteindre plusieurs années. En revanche, sur l’amendement n° II 76, la commission demande l’avis du Gouvernement. Le Président de la République avait annoncé l’acquisition de deux appareils au total. Je sais que le ministère de l’intérieur est en cours de négociation avec la Commission européenne pour l’acquisition d’un appareil dans le cadre d’un financement européen. Toutefois, si les discussions avec la Commission européenne et les constructeurs ont une chance d’aboutir en 2024, ces autorisations d’engagement pourraient sans doute permettre d’accélérer la concrétisation de ces commandes.

que constituent les hélicoptères lourds bombardiers d’eau. La question de l’acquisition de ce type d’appareils doit faire l’objet au préalable d’un travail d’analyse approfondi, eu égard au coût très important et aux conditions de leur utilisation.

ne s’accompagne pas d’un renforcement des moyens de formation de ces jeunes recrues. Les dépenses de formation du programme « Police nationale » étaient de 43,2 millions d’euros en loi de finances pour 2023. Les crédits alloués pour 2024 sont affichés à 29,7 millions d’euros, soit une baisse de 31,5

pour accompagner la politique de recrutement qui est en cours et que nous approuvons. C’est aussi ce que dit la Cour des comptes. Dans son rapport d’exécution budgétaire annuel, le Cour souligne que « pour répondre à l’objectif politique d’un recrutement massif de policiers et de gendarmes, les responsables de programme sont contraints de dégrader la qualité des recrutements et des formations ». La formation des policiers, nous la devons aux policiers eux mêmes, mais également à la population. C’est un levier essentiel de l’efficacité de nos politiques de sécurité publique. C’est pourquoi cet amendement vise à abonder fortement les crédits affectés à la formation des policiers à hauteur de 100 millions d’euros.

En effet, le recrutement au cours de ces dernières années de jeunes policiers ne s’est pas accompagné d’un renforcement suffisant des moyens de formation. L’augmentation du nombre de policiers recrutés devrait s’accompagner du recrutement de nouveaux personnels de formation, afin d’œuvrer pour que notre police nationale soit en pointe, singulièrement dans le domaine des enquêtes, de la lutte contre la criminalité organisée ou la lutte contre les discriminations. Comme nous avons pu le souligner précédemment, ce texte ne prend que peu d’engagements en termes de formation des policiers. Pourtant, pouvoir se former est une demande unanime des forces de l’ordre. Nous sommes convaincus qu’une véritable police du quotidien ne peut pas se limiter à la seule augmentation des effectifs. La formation initiale est trop éloignée des réalités, trop textuelle et trop courte, et la formation continue est pratiquement inexistante. C’est pourquoi notre amendement tend à augmenter les moyens affectés au recrutement de formateurs.

l’augmentation du nombre de policiers recrutés devrait nous obliger à consolider les cycles de formation, en garantissant des moyens importants pour celle ci. Encore une fois, il s’agit d’une demande unanime des forces de l’ordre.

axe, le Beauvau de la sécurité a déjà permis de financer l’augmentation de la durée de la formation initiale et continue des policiers. Vous dites que la formation est trop courte ? La durée des

et de programmation du ministère de l’intérieur sur la période 2024 2027, 118,7 millions d’euros de crédits supplémentaires ont été alloués à la formation. de la présente budgétisation, il est prévu en 2024 11,7 millions d’euros supplémentaires, dont 5 millions d’euros de subventions supplémentaires à l’École nationale supérieure de la police, pour accompagner les besoins de formation induits par l’augmentation du schéma d’emplois. d’emplois. Troisième axe, les structures de formation initiale et continue de la police nationale font régulièrement appel à des formateurs et des intervenants de haut niveau dans les cursus de formation, notamment dans des domaines très techniques en lien avec le cyber ou la préservation et l’exploitation des traces numériques dans les enquêtes.

Les causes en sont multiples : augmentation des coûts du carburant et de l’énergie ou encore multiplication des intempéries, inondations et incendies, ayant pour cause le réchauffement climatique et venant accroître les dépenses d’interventions des Sdis. Alors que les Sdis sont cofinancés par l’État et les départements, ce sont ces derniers qui ont en réalité une place prépondérante dans leur budget de fonctionnement. Les collectivités territoriales, notamment les départements, étant déjà asphyxiées sur le plan financier par la baisse de leurs dotations ces dernières années, nous demandons que l’État assure un concours financier plus prononcé en faveur des Sdis. Tel est le sens de cet amendement, qui vise à abonder les moyens des Sdis à hauteur de 100 millions d’euros.

Tout d’abord, je rappelle que la dotation de l’État pour l’investissement structurant des Sdis a déjà été substantiellement renforcée ces deux dernières années avec la concrétisation des pactes capacitaires.

d’autorisations d’engagement destinée à aider les services d’incendie et de secours à financer l’achat de camions citernes feux de forêt. Or ces autorisations d’engagement résultent d’un amendement gouvernemental adopté à l’Assemblée nationale l’année dernière. Outre 150 millions d’euros en autorisations 37,5 millions d’euros en crédits de paiement pour l’année 2023. Le Gouvernement a procédé de nouveau par amendement cette année, pour inscrire une nouvelle tranche de 39 millions d’euros en crédits de paiement pour 2024. Cette méthode d’action,, pour une mesure annoncée depuis plus d’un an, est profondément insatisfaisante. Elle souffre d’un fort déficit de transparence, contrevient à l’objectif de sincérité budgétaire et constitue un manque de respect flagrant à l’égard du Parlement. Nous n’avons ainsi aucun élément de calendrier relatif à l’engagement des crédits restants, et le projet annuel de performance est lacunaire. Par conséquent, je vous propose, par cet amendement, d’inscrire les 73,5 millions d’euros de crédits de paiement restant à engager. Cette démarche vise, d’une part, à inciter le Gouvernement à anticiper davantage la budgétisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre des pactes capacitaires, y compris dans les documents budgétaires, et, d’autre part, à s’assurer que l’intégralité des autorisations d’engagement votées par le Parlement en 2022 seront consommées. Il y va de la capacité de résilience de nos services d’incendie et de secours.

suppose des investissements constants en maîtrise d’ouvrage. Or, à ce jour, les loyers versés par l’État ne permettent pas de couvrir les besoins de fonctionnement et d’investissement afférents à ces ouvrages. Cette réalité est amplifiée par l’augmentation du coût de l’énergie, des matériaux et des travaux. Le coût réel des investissements à mener est environ le double du coût plafond appliqué qui sert de base pour l’établissement des loyers. Face à une telle conjoncture, dans la perspective d’un déséquilibre financier grandissant, les maîtres d’ouvrage ne peuvent plus engager leur responsabilité dans la reconstruction des gendarmeries existantes. Ainsi, dans la Nièvre, le bailleur social rural Nièvre Habitat se heurte à cette difficulté pour la conduite de quatre opérations de renouvellement du parc de gendarmerie. Les projets sont fortement compromis. C’est pourquoi le présent amendement tend à la création d’un programme nouveau, au sein de la mission « Sécurités », dédié au financement de la rénovation des locaux de gendarmerie et abondé à hauteur de 50 millions d’euros.

Nous proposons en effet d’abonder le programme 152 « Gendarmerie nationale » de 50 millions d’euros pour financer les besoins immobiliers des gendarmeries. De nombreux territoires ont de réels besoins en matière de reconstruction à neuf de leur caserne de gendarmerie. Ces casernes, situées en milieu rural, sont vétustes et ne répondent plus aux normes actuelles de confort et de sécurité, ce qui dégrade nécessairement les conditions de travail et de vie des gendarmes et de leurs familles et met à mal l’attractivité de certains territoires. En outre, le financement des petites casernes soulève des difficultés particulières. Par l’effet du décret du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation des casernes de gendarmerie par les offices

dans le PLF 2024 pour ajuster la subvention d’investissement en collectivité destinée aux petites casernes, en abondant l’action n° 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale

les ministères de l’économie et de la justice, pour intensifier la lutte contre les trafics financiers. Son adoption permettrait de doubler les effectifs de police affectés à la lutte contre la délinquance financière et économique en collaboration avec le fisc, les douanes et la justice financière.

L’année dernière, seuls 34 % des Français ont indiqué avoir suivi une formation certifiante aux gestes de premiers secours. Parallèlement, la subvention aux associations et aux organismes concourant à cette mission de sécurité civile stagne depuis plusieurs années. Nous demandons donc des moyens à la hauteur de ces objectifs. Nous proposons en conséquence d’augmenter ce budget de 10 millions d’euros. Cela permettra une montée en charge progressive de la formation aux gestes de premiers secours, notamment en ciblant prioritairement les professionnels de la petite enfance. Nous demandons par ailleurs au Gouvernement de lever le gage.

sécurité civile » correspond aux activités de coordination et de formation des acteurs de la sécurité civile. Elle comprend également le développement de la résilience de la population au moyen, notamment, de la généralisation de la formation aux gestes de premiers secours.

Les Sdis et les associations agréées de sécurité civile dispensent des formations aux premiers secours, mais ils reçoivent dans ce cadre des ressources propres, puisque ces formations sont facturées. Il ne me semble donc pas opportun d’inscrire des crédits dans le programme 161 pour financer ces formations. Demande de retrait, ou avis défavorable.

Fos sur Mer, Vannes, Carcassonne, Perpignan, Châtel Guyon : de nombreuses écoles de police ont été fermées au cours des dix dernières années.

est l’avis du Gouvernement ? pour augmenter la capacité de formation à court terme. La nécessité d’assurer une formation solide aux policiers constitue déjà une priorité largement financée par le ministère.

comme le précise le document budgétaire de la mission. Ces actions sont financées en dépenses d’intervention à l’action n° 11 du programme 161 « Sécurité civile » à hauteur de 500 000 euros, soit un montant identique à celui de l’année dernière. Alors que cette dépense est stable, il est pour le moins anormal que les dépenses d’intervention du programme diminuent, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement. C’est pourquoi nous proposons d’abonder de 3 millions d’euros les dépenses d’intervention en matière d’actions de prévention des feux de forêt.

Marianne Margaté. Nous nous réjouissons de l’annonce au début du mois de novembre de l’ouverture d’un centre de formation sur la base aérienne de Nîmes Garons. Ce centre formera les futurs pilotes des bombardiers, une flotte de la sécurité civile essentielle à la réalisation des opérations de lutte contre les feux de forêt. Il subsiste pourtant une inquiétude quant au financement du simulateur de vol Dash, d’un coût de 1,5 million d’euros. Or le financement ne peut plus attendre, car nos pilotes doivent se rendre plusieurs semaines au Canada pour apprendre à piloter un tel engin. En outre, le simulateur a vocation à être financé par l’État, et non par les collectivités territoriales. Quel est l’avis de la commission Il me semble que l’acquisition de ce nouveau simulateur est déjà satisfaite par le PLF. Près de 35 millions d’euros sont prévus entre 2024 et 2029 pour le redimensionnement de la base aérienne de Nîmes

qui équipe les Dash d’un système multimissions – feu de forêt et transport –, a prévu l’installation d’un tel simulateur sur la base de Nîmes Garons. Celui ci sera opérationnel pour la fin de l’année 2025. En outre, le coût du simulateur s’élève aux alentours de 20 millions d’euros, Il intègre l’investissement, l’infrastructure et l’environnement nécessaires au fonctionnement du simulateur. Votre amendement ne permettrait donc pas de couvrir

de la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP). Dans le PLF 2024, la participation prévue s’élève à 107 millions d’euros, en hausse de seulement 1,9 % par rapport à l’an dernier. La participation demandée à l’État s’établit, quant à elle, à 110 millions d’euros. Nous déplorons ce décalage assez important entre les crédits demandés et les crédits accordés, en particulier en vue de la conduite des opérations relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques. En cas de sous financement de la BSPP, la seule variable d’ajustement serait celle de la masse salariale, avec pour conséquences un moindre recrutement de jeunes sapeurs pompiers et une dégradation de la réponse opérationnelle de la brigade. C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d’abonder cette participation pour le financement de la BSPP à hauteur de de 1 million d’euros. Quel est l’avis de la commission ? La participation de l’État au budget de la BSPP est une obligation légale et n’a cessé de croître depuis cinq ans, puisqu’elle a augmenté de 18 %.

de la BSPP et dans la perspective des jeux Olympiques 2024, la contribution de l’État au budget de la BSPP est ainsi passée de 88,3 millions d’euros en 2019 à 104,9 millions d’euros en 2023. En 2024, la progression sera de l’ordre de +2 millions par rapport à 2023 pour atteindre près de 107 millions d’euros.

le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, car une augmentation du nombre de psychologues cliniciens est déjà prévue. Le schéma d’emploi adossé à la Lopmi 2023 2027 a déjà acté la création de nouveaux postes de psychologues cliniciens au sein du dispositif d’accompagnement psychologique de la gendarmerie nationale. Ainsi, le nombre de psychologues cliniciens en gendarmerie atteindra 85, contre 43

Elle vise à répondre aux critiques qui sont adressées aux mécanismes actuels de contrôle interne des forces de l’ordre : manque d’indépendance, soupçon de partialité, effet de corps ou encore perte de confiance avec la population. Une telle réforme a déjà été appelée par les ministres. Le Président de la République lui même avait évoqué

aux voix ces crédits, modifiés. Nous allons procéder à l’examen des amendements portant sur les objectifs et indicateurs de performance de la mission « Sécurités », figurant à l’état G.

était l’un des fils rouges du Beauvau de la sécurité. Par ailleurs, les forces de sécurité elles mêmes peuvent être victimes d’actes de discrimination émanant de leurs collègues ou de la population. Par la création de cet indicateur, nous pourrions assurer le suivi de ces actes dans le cadre du PLF.

comme vous le savez, le Gouvernement est pleinement engagé dans la promotion de l’égalité professionnelle et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Ensuite, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure dispose déjà

conformément à l’objectif fixé par le Parlement de rationaliser le volume des indicateurs dans les projets annuels de performances

Il paraît donc légitime que l’institution des forces de sécurité puisse mener elle même ses propres études et statistiques. L’examen de cet amendement est l’occasion de rappeler que la question des contrôles d’identité représente un enjeu central de la qualité du travail de nos forces de sécurité et du lien de confiance avec la population.

dont les policiers et les gendarmes disent eux mêmes qu’ils ont besoin. Cet amendement vise ainsi à mettre en place un indicateur permettant d’évaluer le nombre de jours de formation continue suivis par les policiers et les gendarmes.

nous prévoyons des modalités d’actualisation très favorables du nouveau loyer, puisque la période de vingt sept ans couvre généralement la durée des crédits des propriétaires. Je mets aux voix

de la commission des finances d’examen séparé de certains amendements portant sur les crédits de la mission « Cohésion des territoires », ainsi que d’une demande tendant à faire en sorte que les amendements de la mission « Enseignement scolaire » et de la mission « Recherche et enseignement supérieur » soient classés de façon à permettre des regroupements par thématique.

La séance est levée.